ses ressources tout en continuant d'augmenter ses droits à la retraite. La nécessité de l'accord de l'employeur limite considérablement l'accès au dispositif. L'article 13 encadre le refus de temps partiel de l'employeur, lorsque la quotité de de travail souhaitée est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise. L'appréciation de la compatibilité entre la quotité de travail et des besoins de l'activité économique de l'entreprise rend,, inapplicable l'accès à la retraite progressive. Nous estimons que la retraite progressive doit être, pour les travailleurs, un droit qui s'impose aux employeurs. J'en profite pour saluer l'ensemble des salariés et leurs familles qui ont manifesté, pour certains ce matin

Si nous souscrivons à l'idée d'élargir le bénéfice de la retraite progressive à l'ensemble des assurés, le dispositif est vidé de sa substance par la possibilité laissée à l'employeur de refuser aux salariés

pas seulement la question de l'intensité du travail, mais aussi celle de la liberté de choisir le moment et la manière de partir à la retraite, au regard des conséquences sur le montant de la pension. Le recul de l'âge légal à 64 ans contraint

une retraite insuffisante, soit de s'user davantage au travail. L'aménagement du temps de travail en fin de carrière ne peut être limité par un refus de l'employeur sans explication au salarié. Pour ces raisons, nous demandons que ce refus soit motivé par écrit. Je dis bien, car vous l'aurez compris, toutes nos interventions visent à demander le retrait de cette réforme. À cet égard, nous sommes solidaires des manifestations qui ont lieu partout dans le pays, aujourd'hui encore. Quel est l'avis de la commission

proposé que le Comité national consultatif des personnes handicapées donne son avis avant que le Gouvernement ne prenne un décret sur les conditions de cumul de la pension d'invalidité avec une retraite progressive. Nous avons présenté cet amendement dans le but d'enrichir et de préciser le texte. Cependant, il ne pourra être soumis au vote puisque, comme vous le savez maintenant par coeur, ... vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. D'ailleurs le journal de cet après-midi titre les débats ». Eh bien, nous ne sommes anesthésiés ni par le chloroforme de l'article 47-1 de la Constitution, ni par le 44.2, ni par le 44.3, ni par vos amendements qui n'avaient pour but que de faire tomber nos propres amendements, ni par l'article 38 du règlement du Sénat, ni, enfin, par le 46 . Nous ne lâcherons Nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons pas les Français et nous continuerons à nous battre contre ce projet de réforme des retraites.

La retraite progressive est un dispositif essentiel pour le maintien en emploi des seniors et la prise en compte de l'accroissement de leur vulnérabilité face aux risques psychosociaux en selon les chercheurs Serge Volkoff et Corinne Gaudart, nombre de seniors se maintiennent en activité professionnelle à condition de disposer d'un aménagement du temps de travail qui leur convient. La sortie d'un système contraignant en termes d'horaires ou de rythme est alors, pour ces personnes, une condition pour ne pas sortir de la vie active. Afin de prévenir l'augmentation des risques et de permettre à un maximum de personnes de profiter de la retraite progressive, il est important

avant l'âge d'ouverture des droits -, le présent projet de loi constitue un frein pour de nombreux seniors, qui devront attendre d'avoir 62 ans pour en bénéficier.

est rédigé en corse, j'espère que ma traduction sera fidèle : « Vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre vos mains. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Ils sont dans la rue aujourd'hui. Nous ne lâcherons rien ; nous ne les lâcherons pas. » J'espère, cher Paulu, que ma traduction de ton corse est exacte. Il manque l'accent

Ce refus ne pourra intervenir que lorsque la quotité de travail souhaitée est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise. L'employeur devra adresser son refus aux salariés dans les deux mois. En revanche, le texte ne précise pas que l'employeur doive motiver son refus aux salariés. L'employeur pourrait en conséquence adresser un refus aux salariés sans justifier de l'incompatibilité du temps partiel avec l'activité économique de l'entreprise, voire sans donner aucune justification.

pour vous dire que vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute- nous vous l'avons dit de nombreuses fois ... Ah bon ? ... que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes ; les Français n'ont plus ! Nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons pas, c'est pour cela que je vous présente cet amendement. Le projet de loi encadre les possibilités de refus de temps partiel de l'employeur en cas de demandes de salariés souhaitant bénéficier de la retraite progressive. En vertu des règles introduites, l'employeur ne pourra refuser le temps partiel que lorsque la quotité de travail souhaitée est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise. Il devra adresser son refus au salarié dans les deux mois. Or le projet de loi ne précise pas que l'employeur doive motiver son refus au salarié. L'employeur pourrait en conséquence adresser un refus au salarié sans justifier de l'incompatibilité du temps partiel avec l'activité économique de l'entreprise, voire sans donner de justification.

Selon la Drees, le dispositif de retraite progressive concernait 24 000 personnes en 2020, ce qui est vraiment une honte. Il est, selon les termes mêmes de cette étude, très marginal. Voulons-nous vraiment que plus de personnes puissent bénéficier de la retraite progressive à temps partiel, dispositif vertueux de transition entre l'emploi et la retraite ? Voilà une solution simple

90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et votre seule réponse, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale, et surtout mépris du Président de la République envers les syndicats qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le ! L'amendement

d'éligibilité au dispositif soit porté de 60 à 62 ans, considérant que la retraite progressive doit constituer un outil de prise en compte des carrières pénibles en permettant l'allégement de la charge de travail de l'assuré

comme pour les nouveaux. Si la majorité sénatoriale est favorable au dispositif de retraite progressive, il faut créer les conditions pour permettre son application effective. C'est le sens de notre amendement, à supprimer la possibilité pour l'employeur de refuser la retraite progressive à temps partiel en raison de l'incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. L'amendement

manifestations historiques, 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et votre seule réponse, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le ! Si nous souscrivons à l'idée d'élargir le bénéfice de la retraite progressive à l'ensemble des assurés, le dispositif est vidé de sa substance par la possibilité laissée à l'employeur de refuser aux salariés le bénéfice de la retraite progressive, s'il juge que le temps partiel demandé est incompatible avec l'activité de l'entreprise. Autant dire que pas mal de portes vont se fermer ! Il faudrait au contraire faire du passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive un droit faute de quoi ce dispositif ne bénéficiera qu'à une poignée de salariés- je pense notamment aux cadres, qui sont souvent au forfait. Pour les métiers à forte pénibilité, cette aspiration à la réduction du temps de travail avant d'arriver à la retraite est plus que justifiée.

manifestations historiques, 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et votre seule réponse, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale, et surtout mépris du Président de la République envers les syndicats qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le ! L'amendement que je m'apprête maintenant à défendre et qui a été déposé par le groupe écologiste vise à demander au Gouvernement un rapport- je sais ce que vous pensez de ces demandes -qui présente

emploi-retraite ne bénéficie majoritairement qu'aux personnes qui ont occupé un emploi de cadre, qui sont en bonne santé et qui ont une pension de retraite correcte. Ce qui est prévu ici va précariser encore un peu plus les retraités qui ont de petites pensions et pousser les plus pauvres à travailler au-delà de 64 ans. Encore une fois, la priorité du Gouvernement et de la majorité sénatoriale devrait plutôt être de corriger les inégalités de carrière, qui concernent majoritairement les femmes, et d'augmenter les pensions de retraite, qui sont largement insuffisantes. Cet article montre que, non content de forcer les Françaises et les Français à travailler deux ans de plus, le Gouvernement refuse d'augmenter les pensions et pousse les Français les plus précaires à travailler au-delà de 64 ans. Quel

les modalités ont été précisées par le décret du 31 décembre 2011 relatif à la mise en oeuvre des prestations du droit à l'information des assurés sur la retraite. Ce dispositif permet aux assurés de plus de 45 ans d'obtenir, à leur demande, un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite ou encore sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite. Cependant, la plupart des assurés, en particulier les plus fragiles, ignorent ce droit. Selon une étude basée sur la génération 1968, parmi les affiliés aux régimes de retraite qui ont validé un droit entre 30 et 40 ans, 22 % des femmes ont cotisé moins de dix années à l'âge de 45 ans. Ce pourcentage est moindre pour les hommes- 12 % -, mais il reste préoccupant. Cet amendement tend donc à inverser l'initiative de la rencontre, en imposant aux organismes de retraite de contacter les assurés dont la durée d'assurance est inférieure à dix années et de leur proposer un entretien d'information adapté à leur situation. L'amendement n° 1401, présenté

Nous avons estimé que les dispositions actuelles en ce qui concerne l'information étaient suffisantes, raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable

Venons-en à l'amendement ! Six manifestations historiques, 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et votre seule réponse, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale, et surtout mépris du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, vous devez le retirer ! Par cet amendement, nous voulons attirer l'attention sur la situation des plus anciens, qui n'ont pas toujours accès à internet. Même s'il existe une possibilité de prendre rendez-vous, faut-il encore avoir l'information et le numéro de téléphone, lequel est uniquement disponible sur le site internet ! Vous comprenez, mes chers collègues, monsieur le ministre, la difficulté de nos concitoyens n'ayant jamais utilisé un ordinateur de leur vie pour accéder simplement à des informations sur leurs droits.

pénalise les assurés titulaires d'une retraite anticipée au titre du handicap ou d'une retraite au titre de l'inaptitude au travail, qui bénéficient légitimement d'un régime de faveur et d'une réduction de la durée d'assurance exigée afin de tenir compte de la réalité du marché du travail, de leur fatigabilité et de leurs conditions de travail. travail. Cet amendement vise à permettre aux titulaires d'une pension liquidée au titre de l'inaptitude et aux titulaires d'une retraite anticipée de bénéficier du cumul emploi-retraite intégral. Quel

par un régime de retraite obligatoire français sont toujours en vie. Toutefois, la mise en oeuvre de cette mesure, qui doit permettre de renforcer les moyens de la lutte contre la fraude aux prestations sociales, a été plusieurs fois repoussée ces deux dernières années. À ce jour, le décret d'application

de l'accès aux prestations pour les Français établis à l'étranger. C'est une première brique pour le chantier que nous aurons à mener sur les différentes conventions.

qui partage des valeurs communes. Je crois que la gauche, depuis le début de ce débat, aura donné raison à Camus et illustré ses propos. Surtout, et ce sera ma conclusion,

Encore une mobilisation record ; encore des chiffres records, partout en France ! Six manifestations historiques, 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et votre seule réponse, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris, surtout, du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le ! Comme le chantent en ce moment une partie de nos collègues partis manifester pour exiger le retrait de cette réforme scélérate, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur : « Nous, on est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là

La parole est à M. Daniel Salmon. Afin de prévenir l'augmentation des risques et de permettre à un maximum de personnes de profiter de la retraite progressive, il est important que l'âge d'accès au dispositif corresponde à un âge cohérent avec l'accroissement de la vulnérabilité.

inflation liée au choc énergétique, accélération des conséquences du changement climatique, notamment des canicules, qui ont fait plus de 3 000 morts en 2022 ... Alors que tout s'effondre, le bon sens voudrait que le Gouvernement donne la priorité aux urgences écologiques et sociales résultant de ces bouleversements et anticipe les chocs à venir. À l'inverse, la réforme des retraites proposée illustre l'impensé social et climatique du Gouvernement. Elle est une nouvelle illustration de l'obsession productiviste pour la croissance du PIB, qui mène au chaos, en ignorant les limites planétaires, la souffrance sociale et la perte de sens au travail. Elle est fondée sur l'idéologie de la croissance infinie travailler plus, pour produire plus, pour consommer plus, à contre-courant des besoins de sobriété et de décroissance que nécessite l'urgence climatique. La planète brûle et les droites jugent urgent de reculer le départ à la retraite. Elles ne souhaitent qu'une chose : aggraver encore et encore les injustices sociales. C'est inique et absurde. manifestations historiques, 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et votre seule réponse, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris, surtout, du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le

de retirer. Ce projet mérite toujours d'être transformé. En l'état actuel des choses, comme mon collègue Pierre Ouzoulias le sait, l'ensemble des enseignants-chercheurs,

qui vise à permettre le rachat de trimestres de stage ou d'études pour que les assurés qui ne disposeraient pas du nombre de trimestres requis pour liquider leurs droits à taux plein puissent réduire la décote applicable à leur pension. Afin de garantir l'effectivité de ce dispositif, cet amendement tend à assigner aux établissements d'enseignement un rôle d'information auprès des élèves et des étudiants sur les droits qui leur sont ouverts.

la protection sociale. Cependant, il ne me paraît pas utile de l'inscrire dans la loi. Nous savons que le dispositif de rachat de trimestres a été reculé à l'âge de 30 ans, ce qui laisse le temps nécessaire de la réflexion. Il ne faut pas non plus que ce soit trop long, parce que, plus ça tarde, plus c'est cher.

Poncet Monge. Nous entamons l'examen d'une série d'articles sur les trajectoires de financement des branches de la sécurité sociale, que nous jugeons insincères. Les budgets prévisionnels de la branche maladie ne tiennent pas compte des dépenses induites par l'inflation.

alors que le travail s'intensifie et que les accidents du travail augmentent. Selon le chercheur Nicolas Dufour, le taux d'incidence des accidents mortels et non mortels a augmenté de 47 % en France, en faisant la plus mauvaise élève de l'Union européenne concernant les accidents du travail.

J'espère que la traduction sera fidèle ... Paulu Parigi me dit que, malheureusement, à cause de la tempête, les Corses n'ont pas pu manifester, mais il rappelle qu'ils qu'ils ont participé aux six manifestations historiques précédentes, et qu'ils étaient 9 000 à le faire. Il vous rappelle aussi que 90 % des actifs sont opposés à la retraite à 64 ans, et que la seule réponse ne peut être le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris

peu nombreux et majoritairement situés dans ou autour de Mamoudzou, le chef-lieu, d'importantes zones de l'île, notamment le Nord et le Sud, demeurent très largement sous-dotées.

47 % des plus de 65 ans estiment que leur état de santé est mauvais ou très mauvais. Enfin, l'espérance de vie y est de 75 ans, soit inférieure de huit ans à celle de l'Hexagone. L'amélioration de l'accès aux soins sur le territoire doit représenter une priorité. Celle-ci passe par le développement de l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé. Cet amendement vise ainsi à affilier les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins conventionnés avec l'assurance maladie qui résident et exercent leur activité à Mayotte aux régimes de prestations complémentaires de vieillesse dont bénéficient déjà ces professionnels en métropole. En contrepartie, l'assurance maladie prendra en charge une partie des cotisations des professionnels affiliés. Le bénéfice de ces régimes permettra aux professionnels de santé exerçant à Mayotte d'améliorer significativement leur pension de retraite. Monsieur le ministre, les Mahorais vous savent gré d'accéder à cette demande importante des professions libérales locales. Cette mesure contribuera à lutter contre la désertification médicale et à améliorer sensiblement l'accès aux soins. sur la nécessité d'affilier les professionnels libéraux de la médecine aux régimes complémentaires de pensions de vieillesse, pour redonner de l'attractivité et corriger une inégalité. Le Gouvernement a déposé un amendement strictement identique pour lever le gage et rendre celui de M. le sénateur recevable. Quel est l'avis de

Poncet Monge, sur l'article. L'article 14 est le premier d'une longue série d'articles sur les trajectoires financières des branches de la sécurité sociale. Nous l'avons dit, il nous semble très difficile d'établir la sincérité de ces multiples trajectoires, tant les externalités négatives, notamment sur les autres branches, mais aussi macroéconomiques, sont importantes, sans être prises en compte dans les calculs du Gouvernement.

de la réforme de 1993, en France, sur la santé perçue- aussi bien mentale que physique. Une autre étude, menée par l'université de Jérusalem en 2018, a examiné l'effet d'une réforme comparable, adoptée en Israël en 2014, et montré que celle-ci avait été préjudiciable à la santé. en évoquer d'autres, mais mon temps de parole est contraint. Quoi qu'il en soit, la conclusion est toujours la même : les réformes des retraites, notamment des paramètres que vous privilégiez, en particulier celui de l'âge, dégradent la santé, car elles obligent à travailler plus longtemps, alors que l'on observe une intensification du travail, que tous les facteurs de pénibilité explosent et que le management néolibéral a des effets délétères, voire toxiques- je vous renvoie à France Télécom ! La parole

Mépris envers l'opposition sénatoriale, ce qui n'est pas le plus grave. Mépris, surtout, du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet est illégitime, nous vous demandons de le retirer

de l'usure professionnelle, dont le coût est estimé à 30 millions d'euros pour l'année en cours. Je ne peux que regretter que nous n'ayons pu discuter de ce fonds lors de l'examen de la négation de notre rôle par le Gouvernement, avec le recours à l'article 44.3 de la Constitution, nous n'avons pas pu défendre ces travailleurs de la fonction publique hospitalière, dont le métier, très exigeant, usant, pénible, méritait plus de reconnaissance. pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), beaucoup de soignants tirent encore et toujours la sonnette d'alarme. En effet, ces travailleurs, dont la charge de travail ne cesse de s'accroître face aux pénuries de personnel dans les hôpitaux, subiront de plein fouet le recul de l'âge de la retraite. Pour ces métiers, la prévention et l'aménagement de la fin de carrière requéraient, au minimum, un plan de soutien d'envergure ; ce que vous proposez est dérisoire au regard des besoins. Il est grand temps de prendre la mesure des difficultés de notre système hospitalier et de la souffrance de ses personnels et d'y apporter une réponse ambitieuse santé de nos concitoyens. Il nous faudrait nous réjouir des 750 millions d'euros de rallonge budgétaire. Mais il manque bien plus que 750 millions d'euros pour notre système de santé, hôpital et médecine de ville Il faut redonner aux agents de l'hôpital la capacité de faire leur métier. La vérité financière de la branche maladie, c'est que les cotisations sociales, salariales et non salariales, ne représentent plus que 36 % des financements. Il suffit de lire la page 36 de l'annexe 3 du PLFSS 2023 pour s'en convaincre. Les cotisations sociales seraient encore freinées par le dynamisme attendu des allègements généraux, mais aussi par la baisse des cotisations maladie des travailleurs

Pis, la branche maladie peut leur apparaître comme injuste, car elle est financée davantage par la TVA et par la CSG, pour 129,3 milliards d'euros. Avec ce type de recettes, les ministres se relaieront pour dire que ce n'est pas possible ou, comme aujourd'hui, pour venir présenter les miettes consenties au monde de la santé. Rien qu'en ce début d'après-midi, 257 amendements sont tombés en une seconde. Six manifestations historiques, 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et votre seule réponse, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris, surtout, du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir.

vous me direz : à quoi bon, puisque vous-mêmes dévitalisez la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures offertes par la Constitution et par le règlement

». Nous l'avons remarqué, avec le refus du Président de la République de recevoir l'intersyndicale, avec, depuis le départ, le refus de négocier vraiment cette réforme, et, aujourd'hui, le passage en force au Parlement.

L'arbre tient bon ; le roseau plie. « Le vent redouble ses efforts, « Et fait si bien qu'il déracine « Celui de qui la tête au ciel était voisine, « Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Je veux saluer les Français qui travaillent, qui font tourner le pays, qui manifestent aujourd'hui, qui ont voté contre l'extrême droite et qui vous permettent, monsieur le ministre, d'être assis au banc du Gouvernement, alors que vous n'avez pas de vraie majorité à l'Assemblée Je veux saluer les Français qui se battent pour défendre leurs droits, et dire que nous ne les lâcherons pas

90 % des actifs qui sont opposés à la retraite à 64 ans, et la seule réponse du Gouvernement, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Surtout, et bien plus grave, mépris du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le ! Avec cet amendement, qui vise à supprimer l'article 14,

cette réforme. Allez-vous finir par les entendre, au-delà de ce que nous vous répétons chaque jour dans cet hémicycle ? Je vous le demande, monsieur le ministre : entendez-les ! Dites au Président de la République de les entendre et retirez votre réforme

par ce qui s'apparente à un aveu de faiblesse, vous nous privez de la discussion sur ce sujet important, qui concerne la santé de nos concitoyens. De fait, vous avez anesthésié les débats. C'est bien dommage. Les Français attendaient nos débats et comptaient sur nos propositions pour vous faire abandonner cette réforme, qu'ils considèrent comme néfaste pour eux. Pour quel résultat ? Six manifestations historiques, 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et une seule réponse de votre part : le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris, surtout, du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Mépris, enfin, envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le

à pleine cotisation est censé être de 1 600 euros- sur un mois de départ en 2021, 12 % en décote pour incapacité de travail et 24,5 % en décote. Alors que le montant théorique de pension complète de cotisations est de 1 600 euros, le montant réel moyen de la pension de départ à la retraite est de 1 000 euros, d'après un rapport de l'assurance retraite allemande datant de 2022. Le taux de pauvreté monétaire en Allemagne est le triple de celui de la France, d'après les chiffres de l'OCDE en 2019. Ainsi, 7,85 % des femmes allemandes sont en dessous de 1 200 euros, et 60 % sous les 900 euros. Le système allemand est particulièrement brutal pour les femmes. Voilà donc le modèle qui vous inspire pour votre réforme ! Il est profondément injuste et brutal. C'est pourquoi, comme les milliers et milliers de personnes qui sont dans la rue aujourd'hui, nous vous demandons de nouveau de retirer cette réforme. La parole est à Mme Annie

ne nous permet pas d'en discuter, nous en demandons la suppression. Le plafond proposé est certes en augmentation- +3,6 % par rapport à 2022 -, mais à un niveau largement inférieur à celui de l'inflation, prévu est de 4,3 %. Cela représente ni plus ni moins qu'une baisse des dépenses qui couvrent les risques maladie, maternité et invalidité. Sans grande surprise, aucun des objectifs fixés n'est à la hauteur nos besoins. Les Français vous le disent : six manifestations historiques, 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et la seule réponse, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris, surtout, du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le ! Tout au long du débat, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, avec les autres groupes de gauche, s'est attaché à le dire : l'urgence, ce n'est pas la réforme des retraites, mais un financement massif

Plus de 6 millions de Français, dont 600 000 sont atteints d'une affection de longue durée, n'ont pas de médecin traitant. Ces chiffres sont très inquiétants. La désignation d'un médecin traitant est souvent difficile, voire impossible pour des personnes habitant des zones sous-denses.

dédié au déploiement de politiques de prévention de l'usure professionnelle et d'aménagement des fins de carrières dans la fonction publique hospitalière, et plus particulièrement pour les professionnels de santé employés dans des structures publiques sanitaires et médico-sociales. Son coût est estimé, pour l'année 2023, à 30 millions d'euros. Le secteur sanitaire et médico-social fait face à une à une pénurie de bras. Les métiers de ce secteur sont en grande difficulté et les professionnels se sentent méprisés. Alors que la pénibilité au travail aurait dû être un sujet central de ce projet de loi, votre gouvernement n'y a consacré qu'un seul article. De plus, ce fonds évoque l'usure professionnelle, car vous refusez toujours de parler de pénibilité. Ce choix sémantique souligne la méconnaissance du labeur enduré par des millions de salariés. Vous avez beau bannir de votre vocabulaire le terme de pénibilité, vous n'effacerez pas ses conséquences pour les salariés. Le Président de la République et la droite sénatoriale veulent que les Français travaillent plus longtemps. Mais pour travailler plus longtemps, il faut déjà pouvoir travailler. Ce fonds est très insuffisant. Son montant relève du mépris. Au reste, il est vrai que les salariés du secteur sanitaire et médico-social sont habitués au mépris du Gouvernement.

Comme vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition et le recours à toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement et comme le Président de la République vient désormais de nier le concept même de démocratie sociale, vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées, dont vous faites évidemment partie. Cela a déjà été dit ! Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus ; nous ne les lâcherons pas, nous ne lâcherons rien.

C'est une profonde injustice et c'est une insulte faite à tous ceux qui ont commencé à travailler tôt, à tous ceux qui ont des métiers éreintants et, surtout, c'est une insulte à toutes les femmes, qui seront les grandes perdantes de cette réforme.

à ces âges, 44 % des Français n'ont pas de travail et se retrouvent dans une grande précarité. « Voilà pourquoi je n'ai pas voté l'article 7 sur le report de l'âge légal. « Oui je suis de droite, »- vous l'êtes également -« mais cette réforme n'est pas la mienne. Que M. Macron et son gouvernement l'assument seuls. » Vous devriez méditer ces propos.

le vent se lève, il est temps de vivre, mais il est surtout urgent d'écouter ! Avec cette réforme, le Président de la République joue les apprentis sorciers. Au reste, nous ne sommes pas surpris

de surdité, Merlin risque de casser sa baguette, et Jupiter de voir la foudre se retourner contre lui. Faute d'écouter le peuple qui gronde, nous invitons ceux qui sont dans cet hémicycle à entendre la colère sourde, mais puissante, qui s'exprime chez les Français : six manifestations historiques, 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et votre seule réponse, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris, surtout, du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le ! Après avoir refusé la concertation au au mépris de la démocratie sociale, après le dévoiement de la procédure parlementaire, voilà désormais le passage en force tous azimuts dans les deux chambres du Parlement. Il n'est pas trop tard, retirez ce projet

votre seule réponse, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris du Président de la République envers les syndicats. Mépris envers les salariés et les Français. Retirez votre projet !

malgré le fait que vous ayez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées.

qui est plus un oukase de Bercy qu'un texte de progrès social, qui répondrait aux défaillances et aux déficiences de notre système de santé. Aussi, en cohérence, nous rejetons la rectification de l'objectif de la branche maladie, maternité, invalidité et décès que propose le Gouvernement au travers de cet article.

La justice sociale ne peut jamais fonctionner à l'envers. Nos concitoyens comprennent parfaitement qu'on leur fait payer un impôt sur leur vie,

et votre seule réponse, c'est le mépris : mépris envers l'opposition sénatoriale, car, faisant preuve d'un courage extraordinaire, vous venez de faire tomber 257 amendements que nous aurions pu examiner ensemble

tient compte de l'inflation et de la croissance démographique. Vous imposez une nouvelle cure d'austérité aux régimes sociaux, au mépris de la santé des Français. Pourtant, notre système de santé est déjà en souffrance. Alors que la pandémie du covid-19 a mis en exergue l'extrême fragilité de notre système sanitaire et social, la menace de fermeture de maternités,

auxquels nos compatriotes sont très attachés. Ils vous le disent encore aujourd'hui en manifestant massivement contre vos réformes et nous vous le disons, en continuant de faire notre travail de parlementaire alors que celui-ci est méprisé, tout autant

mépris. Mépris envers nous, l'opposition sénatoriale, puisque nous ne pouvons ni voter nos amendements ni prononcer d'explications de vote. Mépris du Président de la République envers les syndicats,

dont la mécanique de recul de l'âge légal de départ était tout à fait similaire à celle dont nous discutons. Les conclusions de cette étude sont formelles

votre seule réponse est encore le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris du Président de la République envers les syndicats, qu'il ne daigne pas recevoir. Mépris envers l'ensemble des salariés et des Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le

Je ne reviendrai pas sur les conclusions du COR qui battent en brèche votre discours alarmiste sur l'impérieuse nécessité de mettre en oeuvre cette réforme ni sur les efforts que votre gouvernement attend des Français les plus modestes pour réaliser des économies, tandis que les aides et les cadeaux fiscaux aux entreprises ne cessent de croître. Vous faites peser la charge de votre réforme sur la classe sociale

qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le

de la refondation, ce serait une erreur dramatique. Le principe en est simple : toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a le droit à une prise en charge de ses frais de santé de manière continue, tout au long de sa vie. Nous avons amélioré d'année en année, de réforme progressiste en réforme progressiste. Aussi, je me demande sur quoi se fonde le Gouvernement pour prévoir une augmentation de dépenses à hauteur de 100 millions d'euros.

comme une flèche portée contre ceux qui donnent tout et n'attendaient pas grand-chose sinon qu'on les respecte,

à 64 ans. Et votre seule réponse, c'est le mépris : le mépris envers l'opposition sénatoriale et, surtout, le mépris du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Ce projet n'est pas légitime.

Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. « Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. » J'imagine que tout le monde

Inversement, toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme ». Voyez-vous, monsieur le ministre, vous nous faites très peur, votre mépris nous inquiète. Vous pouvez encore retirer ce projet

En guise de rectification de cet objectif, le Gouvernement nous propose un chiffre qui ne tient pas compte d'un certain nombre de réalités : de l'inflation, bien sûr, mais aussi de la croissance démographique ou encore de la progression des maladies chroniques. L'objectif de dépenses proposé est donc largement insuffisant pour répondre aux grands défis auxquels nous faisons face. L'inquiétante détérioration de l'hôpital public, qui s'accélère désormais de mois en mois, ne sera pas contenue et encore moins réparée. Cette crise de l'hôpital s'est

motivera les futures générations. Déjà 10 % des étudiants en médecine abandonnent leurs études en cours et 20 % des places en deuxième année de formation de sages-femmes ne sont pas remplies. J'avais proposé un amendement visant à prendre en compte les stages obligatoires réalisés dans le cadre de la formation de sage-femme pour le calcul de la retraite, comme piste pour revaloriser cette filière, mais nous

et l'opposition sénatoriale, mais surtout le mépris du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir, et envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime

Ce mépris envers les salariés et les Français est inadmissible. Votre projet n'est pas légitime, il faut le retirer.

très petites mesures positives feront passer la pilule du report de l'âge de la retraite à 64 ans. Pas du tout ! Nous abordons l'examen de l'article 14, qui entérine les objectifs de dépense de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour 2023.

évidemment, on peut saluer les rallonges, mais il faut tout de même préciser que les hôpitaux ne peuvent tenir sur des rallonges octroyées de façon discrétionnaire et sans vision pluriannuelle.

dans les métiers du soin, sur les démissions en cascade, sur la crise que vivent les soignants. Les rallonges ne pourront jamais se substituer à une réelle vision de la politique de santé, à un engagement de l'État dans la durée en faveur de notre système de soins et des soignants qui tiennent notre pays.

Voici aujourd'hui la réponse en acte : aucune ambition pour notre hôpital. Je le répète, il nous faut un plan Marshall pour l'hôpital, à moins que votre véritable volonté

90 % des actifs sont opposés à la retraite à 64 ans et votre seule réponse est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le

puisque vous avez utilisé tous les actes de procédure possible pour dévitaliser la fonction parlementaire, nous sommes contraints de présenter des amendements de suppression, non pas pour demander moins, mais pour demander plus en faveur de l'hôpital public. Vous vous rendez compte des conséquences de la politique que vous menez depuis 2017 et qui était censée faire bénéficier les Français du « ruissellement » qu'aurait entraîné la politique de l'offre :

absurdes, mais il n'est pas absurde de continuer d'interpeller le Gouvernement, pour qu'il retire son projet de loi, et nos collègues de la majorité sénatoriale, pour qu'ils ne le votent pas.

» ? Depuis de nombreuses semaines, six manifestations historiques se sont déroulées, dont une cet après-midi, 90 % des actifs sont opposés à la retraite à 64 ans et votre seule réponse, c'est le mépris.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous avez décidé d'utiliser tous les moyens offerts par le règlement du Sénat et par la Constitution pour nous faire taire, car vous n'imaginiez pas que les travées de gauche vous opposeraient pied à pied des arguments construits, cohérents et correspondant à l'intime conviction des Français, qui considèrent, comme nous, que votre réforme est injuste et inutile. Vous vouliez nous faire taire parce que, au fur et à mesure de nos propositions, vous vous trouviez de plus en plus gênés aux entournures et parce que des fissures apparaissaient et s'élargissaient au sein de votre prétendue unité. Vous avez choisi cette facilité sans même imaginer qu'elle représenterait un véritable aveu de faiblesse. Votre attitude provoque mon inquiétude. Comment allez-vous répondre devant les Français, que vous représentez, des basses manoeuvres que vous avez organisées dans cet hémicycle ? Plus sérieusement, je m'inquiète de l'atterrissage de cet épisode au Sénat et de ses conséquences pour notre République. Chacun comprendra

Cette loterie qui donnerait aux travailleurs ayant commencé avant 21 ans un traitement différent selon leur âge en début de carrière est ubuesque. Personne ne peut ni l'expliquer sérieusement ni le justifier politiquement. La cohérence et la justice dans le traitement des Français ne sont pas un détail, c'est une exigence fondamentale, qui conditionne l'adhésion des travailleurs à une réforme et au pacte social.

sous-objectifs. Il confirme la baisse des dépenses de santé imposée par le Gouvernement à l'automne dernier. L'Ondam est largement sous-évalué. Lors de l'adoption du budget de la sécurité sociale pour 2023, nous avons déjà fortement critiqué cette baisse de 1,2 % des dépenses de santé par rapport à 2022, tandis que l'inflation s'élève à 4,3 %. L'hôpital public craque de tous les côtés, cela a été dit. Le manque de personnel a entraîné la fermeture de près de 20 % des lits hospitaliers.

Bien entendu, cela nécessite des moyens. C'est parce que nous avons fait le constat que l'hôpital public manquait de moyens et de soignants que nous avions déposé cette proposition de loi. Le relèvement des dépenses de santé consacrées à l'hôpital et à la médecine publics est absolument indispensable. Le Gouvernement évoque souvent la prévention, mais comment faire de la prévention sans soignants ? Comment attirer les soignants et les médecins

L'un d'eux, qui a également voté contre l'article 7, a publié le texte suivant : « Après le 49.3, le 44.3 permet au Gouvernement, certes en toute légalité, de piétiner les débats parlementaires.

de la colère dans les territoires, chez les élus, chez les habitants. Finalement, les seuls bons comptes dans la période, ce sont ceux que font certains élus extrémistes, qui voient leur capital prospérer. Or, sur ces élus, la République ne peut pas compter

mesure le taux de rejet de cette réforme. Entendez-le ! Redevenez un coriace

ce qu'il vient de se passer. Eh bien non ! Je crois que quelque chose a été cassé cette semaine dans la chambre haute et que cela laissera des traces encore longtemps. Ce n'est pas le style de la maison de ne pas écouter, de ne pas rechercher le consensus,

de repartir de l'essentiel, à savoir les besoins en santé du pays. La pénurie de soignants à laquelle notre pays est confronté doit nous interpeller sur la nécessité de rendre

tous modes d'exercice confondus, l'Hexagone compte en moyenne 336,5 soignants pour 10 000 habitants. À titre de comparaison, la moyenne en Europe de l'Ouest est de 407 soignants pour 10 000 habitants. Nous faisons figure de mauvais élèves en termes de densité en infirmiers- nous en comptons 87,7 pour 10 000

est en très nette baisse, alors que nous connaissons tous les immenses difficultés de nos hôpitaux publics- manque de personnel et de moyens en général. Face aux grands défis du futur, vous continuez de tuer à petit feu l'hôpital public.

? Alors que les métiers du soin sont de moins de moins attractifs, vous proposez au personnel de travailler deux ans de plus. Vous avez oublié que vous les avez applaudis ; aujourd'hui, vous les méprisez. Ce n'est que du mépris

au chômage ou en emploi ont des risques accrus de fatigue. Nous avons parlé hier de pénibilité, d'usure professionnelle, de santé au travail.

que nos débats. Le 6 mars 1836, le trappeur Davy Crokett et d'autres- ils étaient 187 - sont tombés face à 5 000 soldats mexicains alors qu'ils défendaient l'autonomie et l'indépendance du Texas.

C'était un projet pour les femmes ! Remarquez, maintenant que j'ai entendu M. Ciotti nous expliquer que le féminisme était une valeur de droite et que cette réforme était de gauche, je prends avec beaucoup de prudence ce que disent les uns et les autres

Il table en effet sur des dépenses d'assurance maladie en baisse, alors même qu'elles s'inscrivent dans un contexte d'inflation de plus de 4 %. Ne pouvant corriger ce chiffre, sous peine de tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution, qui nous interdit la création de toute charge publique, nous proposons la suppression de cet article. À défaut, défaut, il faudra que quelqu'un nous explique par quel miracle les dépenses d'assurance maladie seraient suspendues hors du temps et échapperaient à l'inflation. Or personne, nous le savons, ne nous expliquera rien, puisque le recours du Gouvernement à l'article 44, alinéa 3, nous interdit tout débat sur nos amendements. Nous voilà constitutionnellement réduits à nous exprimer dans le désert.

Vous auriez fait gagner du temps à nos collègues de droite, qui avaient visiblement mieux à faire que prendre douze journées pour décider, en pleine connaissance de cause, que nos concitoyens devront travailler deux ans de plus. Certains d'entre vous ont eu l'indécence de traiter de fainéants les travailleurs attachés à prendre leur retraite à 62 ans.

de financer les établissements de santé à la hauteur des besoins, soit 1,2 milliard d'euros supplémentaire dès maintenant, en suivant une logique des besoins des territoires de santé et non une logique austéritaire à peine atténuée par des rallonges ponctuelles et insuffisantes. Ainsi, la rectification partielle de l'Ondam pour 2022 ne suffit pas à masquer un Ondam pour 2023 qui ne rattrape pas le retard des budgets précédents, d'autant que l'inflation persiste et pèse sur les investissements. Mais, au-delà de cet amendement, cette réforme des retraites pose un débat de fond : quel monde voulons-nous ? Voulons-nous de ce monde qui glorifie la valeur travail, mais qui crée du chômage et de l'exclusion, qui détruit la planète, qui fait pression sur la puissance publique pour l'appauvrir, qui organise la concurrence et l'injustice fiscale ? Plutôt qu'un monde de régression sociale et de désolation environnementale, allons vers plus de commun et de solidarité et construisons un autre héritage, où le travail aurait plus de sens, serait moins pénible et remis à sa juste place. C'est pour inventer cet autre monde et défendre leur retraite que les Français ont participé en masse à six manifestations historiques et que 90 % des actifs sont opposés à la retraite à 64 ans. Votre seule réponse, c'est le mépris. Mépris envers l'opposition sénatoriale. Mépris, surtout, du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir. Mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime, retirez-le ! », demandent tous ceux qui travaillent à l'hôpital et qui travaillent pour nous. La l'amendement n° 4059 rectifié. Nous proposons de supprimer cet article pour vous dire une fois de plus que nous ne pouvons accepter la limitation des dépenses qui en découle, d'autant que d'autres solutions étaient possibles. Monsieur le ministre, vous avez, de manière assez irrespectueuse, utilisé dans le débat national le nom de notre amie Yolanda Díaz, la ministre du travail espagnole. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une négociation, sous pression de la Commission européenne, avec le gouvernement espagnol sur le mode de calcul des pensions de retraite. Or il se trouve que le gouvernement espagnol a, lui, décidé de mettre davantage à contribution les revenus les plus élevés. Le mécanisme finalement retenu a prévu d'accroître l'assiette de cotisations, c'est-à-dire la part du salaire sur laquelle les employés cotisent, pour dégager des recettes supplémentaires. Ce gouvernement a entériné un doublement d'ici à 2029 du taux de contribution au mécanisme d'équité intergénérationnelle qui alimente le fonds de réserve. Tout cela fait partie de propositions que nous avons faites pendant le débat, mais qu'évidemment vous avez toutes écartées. Je crois que les Français ne sont pas dupes des arguments que vous avez tenté d'employer pour justifier votre réforme. C'est exactement pour cela que nous en sommes aujourd'hui à la sixième manifestation historique. C'est pour cela que 90 % des actifs restent opposés à la retraite à 64 ans. C'est pour cela qu'ils ne comprennent pas que votre seule réponse soit le mépris mépris envers l'opposition sénatoriale, mépris du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir, mépris envers les Français et les salariés qui manifestent aujourd'hui. Votre projet n'avait pas de légitimité en entrant dans cet hémicycle ; il en aura encore moins en en sortant après l'utilisation du 49.3 sénatorial. Vous n'avez qu'une seule solution, monsieur le ministre : retirez votre projet

présenterai dans un instant un amendement pour rehausser le niveau de l'Ondam à hauteur de 750 millions d'euros, dont 600 millions au profit des établissements de santé, ce qui permettra de financer la prolongation des mesures d'urgence sur la rémunération du temps de travail de nuit. Nous financerons cette

croissance de l'Ondam sera donc de 3,5 %, hors dépenses de crise, pour faire suite à des annonces de revalorisation salariale pour les personnels des établissements de santé et médico-sociaux, ainsi qu'à des compensations d'inflation- cela a été vu par les différents services de la manière la plus juste qui soit.

la réalité est plus dramatique que cela : 25 % des Français les plus défavorisés sont décédés à 60 ans. C'est non pas la question d'âge qui est importante, mais celle du revenu. M. Assouline a rappelé le niveau de revenu à partir duquel on appartenait aux 5 % des Français les plus favorisés.

ne sont malheureusement pas concernées par ces âges de départ du fait de leur très grande précarité. Le vote est

Est-ce vraiment un propos acceptable dans notre hémicycle ? Est-ce la seule chose que nous aurions à dire aux plus jeunes sénateurs ?

Nous avons tous été jeunes. Je suis prêt à retirer mes propos si notre collègue s'engage à ne plus dire de sottises de la sorte. Mes chers collègues, je vous rappelle qu'en application de l'article 36, alinéa 10, du règlement, les interpellations de collègue à collègue sont interdites, et elles ont été nombreuses depuis quelques jours

vise à préciser les critères sur lesquels reposent les coefficients géographiques. À la Guadeloupe et aux quatre coins du monde, les accentuer. Six manifestations historiques, 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et votre seule réponse est le mépris mépris envers l'opposition sénatoriale, et surtout mépris du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir, mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime ; retirez-le ! Il y aura encore La crise sanitaire a mis en en lumière les difficultés structurelles de l'offre de soins en outre-mer et la sous-dotation généralisée des établissements de santé de ces territoires. Depuis plusieurs années, Mme Jasmin et ses collègues des alertent le Gouvernement sur l'urgence de revoir le financement de ces établissements, notamment par la revalorisation des coefficients géographiques. Dans tous les départements d'outre-mer, les hôpitaux font face à des surcoûts liés à l'insularité, aux dépenses de personnel, aux frais d'approche, de transport et aux taxes, aux évacuations sanitaires, mais également également à la mise aux normes des bâtiments en matière sismique et cyclonique. Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la sécurité sociale aux tarifs nationaux, au forfait annuel et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l'Hexagone, ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux. Quel

Le report de l'âge de départ à la retraite va provoquer, vous le savez, des arrêts maladie de longue durée, des maladies professionnelles et des douleurs et maladies chroniques.

58 % des morts par accidents du travail ont plus de 50 ans, une surreprésentation que l'on retrouve aussi dans les incapacités permanentes liées au travail qui concernent 41 % de cette La fréquence des accidents mortels croît avec l'âge : les salariés âgés de 60 ans ou plus enregistrent le risque le plus élevé, avec 54,2 accidents par milliard d'heures rémunérées. Nous sommes vraiment sur ce plan un mauvais exemple cette réforme n'est pas nécessaire, mais elle est dangereuse pour la santé et la qualité de vie des seniors

tel qu'il avait été adopté à l'automne 2022. Alors que les accidents du travail ne cessent d'augmenter, que la santé mentale des travailleurs se dégrade et que la pénibilité demande de vrais moyens, le Gouvernement maintient un budget stable.

elle aussi, besoin de soutien financier. Par ailleurs, en proposant une diminution des cotisations des entreprises, vous fragilisez à terme cette branche, et vous déresponsabilisez même les entreprises. Je rappelle que la branche AT-MP est financée à 97 % par les entreprises.

ce sont des femmes et des hommes déjà usés à 62 ans qui devront travailler deux ans de plus ; ce sont des femmes et des hommes plus nombreux qui seront en invalidité, car confrontés longtemps, plus longtemps, à la pénibilité. D'autant que votre gouvernement a retiré quatre des dix critères

l'amendement n° 304. Après les excellents arguments de nos trois collègues sur l'article 16, je suis le premier à présenter un amendement de suppression de cet article, qui n'enlèvera rien à personne puisque l'objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles reste stable et qu'il est même en légère diminution dans ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

moins mal que si c'était pire ... Je le dis sans plaisanter, alors que dans notre pays les accidents du travail restent extrêmement nombreux et que le recul de l'âge de la retraite aura des conséquences importantes en matière de maladies professionnelles. Même si nous approchons de la fin de notre débat, même si vous avez voulu- et nous ne cesserons de le répéter -dévitaliser la fonction parlementaire par des procédures destinées

La pénibilité porte sur le travail et sur ses conditions, soit sur une responsabilité collective ; l'usure porte sur les corps des travailleurs, soit sur une responsabilité individuelle. Nous n'avons pas les mêmes valeurs.

l'amendement n° 561. Oui, le travail peut abîmer et l'objectif de dépenses de la branche AT-MP proposé par le Gouvernement s'avère totalement inadapté aux besoins, notamment avec le recul de deux ans de l'âge de la retraite. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article, dont nous aurions aimé débattre. Hélas, votre attitude à l'égard des oppositions de cet hémicycle nous prive du travail parlementaire qui est le nôtre. Vous ne sortirez pas grandis après ce tour de force. D'ailleurs, la rue gronde. Aux six manifestations historiques et aux 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, vous répondez par le mépris. Les Français s'en souviendront

n° 690. L'article 16 maintient la baisse de 2 % en valeur réelle des dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Pour en revenir à l'article 16, en fonction de leur situation, les salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé, d'indemnités journalières et d'une rente pour eux-mêmes en cas d'incapacité permanente ou pour les ayants droit en cas de décès. La branche AT-MP finance aussi des actions de prévention auprès des entreprises. Son excédent pourrait atteindre 2,2 milliards d'euros pour 2023, montant qui viendrait s'ajouter aux 6 milliards d'euros actuels. Cette branche

de la branche retraite par une diminution des cotisations sociales patronales de la branche AT-MP, alors que les besoins sont immenses.

Cette réforme des retraites aura des conséquences sur les AT-MP. Écoutez les Français, retirez cette réforme injuste. L'amendement " Sergent ! interroge Camember, et la terre du trou ?- Que vous êtes donc plus hermétiquement bouché qu'une bouteille de limonade, sapeur ! Creusez un autre trou !- C'est vrai ! " approuve Camember. La simplicité du sapeur Camember, que vous avez reconnu, est alors dépassée en sottise par son supérieur, le sergent Bitur, qui le traite de « double mulet cornu » et lui reproche de ne pas avoir fait le deuxième trou assez grand pour qu'on puisse y mettre la terre qui en a été C'est exactement ce que le Gouvernement est en train de faire au travers de ce projet de loi. Nous assisterons, à partir de 2024, à un transfert de cotisations au profit de la branche vieillesse en provenance de la branche AT-MP

Voilà pourquoi le Gouvernement se comporte comme le sapeur Camember. Voilà pourquoi nous voulons la suppression de cet article. l'amendement n° 885. Je ne vous parlerai pas de trous, mais de vases communicants. Si nous voulons rejeter la confirmation de l'objectif de dépenses de la branche AT-MP proposée par le Gouvernement, c'est que tout est lié dans cette réforme.

suivant : « Je ne vote pas pour votre parti, mais je tenais tout de même à vous remercier d'avoir voté contre le report de l'âge de la retraite à 64 ans. Au vu des votes des sénateurs de droite, c'en est fini pour moi des votes obstacle au RN. Je me rallie donc désormais à ces gens qui n'en peuvent plus. Merci infiniment quand même d'avoir voté contre cet article 7.

conneries » ... Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rejeter la confirmation de l'objectif de dépenses de la branche AT-MP telle que proposée par le Gouvernement dans cet article. Alors que les accidents du travail font 1 000 morts par an, que la santé mentale des travailleurs se dégrade et que la lutte contre la pénibilité exige de vrais moyens, le Gouvernement souhaite maintenir un budget stable pour les accidents du travail et maladies professionnelles par rapport à 2022, sans aucune ambition nouvelle.

... J'ai l'impression, quatre ans après, que les choses ne se sont guère améliorées. Lors des auditions organisées par la commission des de loi, nous avons entendu les représentants du Medef assurer qu'ils étaient prêts à faire quelques efforts- pas beaucoup ! -à condition qu'on les soulage de certaines cotisations sociales. En clair,

souvent commencée jeune, nous avons rappelé combien la prévention était l'angle mort de votre vision du travail au XXI siècle et combien nous étions opposés à vos modalités de prise en compte de la pénibilité dans le calcul des droits à la retraite. L'ambition, la vraie, aurait été de donner une place centrale à la prévention, en rapport direct avec les critères de pénibilité élargis à des situations d'affection sanitaire que vous ne voulez pas voir ni prendre en compte.

Le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 65 à 60 ans en 1983, une revendication de l'union de la gauche depuis les années 1970, était la réponse politique, juridique et ouvrière à la pénibilité du travail.

le nombre de morts dus aux accidents demeure trop élevé en France par rapport à nos voisins, ce qui démontre que nous avons encore à faire.

Beaucoup n'ont pas la chance de travailler dans une entreprise où rivalisent les ressorts de la qualité de vie au travail, un concept qui reste totalement étranger à des pans entiers de notre économie et de nos salariés. Ce terrain doit continuer à être investi. Nous nous étions préparés en ce sens ; vous nous en avez privés, puisque nous savons que tout ce que nous suggérons sera rejeté. Nous demandons toutefois la suppression de cet article, parce que les travailleuses et les travailleurs en France méritent beaucoup mieux que ce que vous proposez.

contre 18 jours pour les moins de 18 ans. Ce phénomène sera mécaniquement amené à augmenter avec le recul de l'âge de départ. Il est donc évident que la branche accidents du travail et maladies professionnelles mériterait davantage de volontarisme de la part du Gouvernement.

dans le secteur des soins aux personnes âgées, retourner une personne alitée pour réaliser une toilette, à domicile ou en Ehpad, est fatigant au quotidien. Cette pénibilité n'est pas reconnue. Elle est parfois handicapante à la longue et très rarement indemnisée. Cela conduit à des arrêts de travail, à des carrières hachées et à des pensions minimes.

La branche accidents du travail et maladies professionnelles regroupe la prévention à la réduction des risques professionnels, la reconnaissance des sinistres, l'indemnisation des victimes, etc. Elle est donc très importante. L'impératif d'équilibre financier, que vous nous avez confirmé,

des femmes des services à la personne sont deux à trois fois plus longs que les arrêts maladie des salariés du BTP. Il y a donc là un sujet spécifique, si l'on veut réellement

à quel point notre pays a besoin d'autres réponses. De manière extrêmement responsable, nous avons très majoritairement, dans les rangs de la gauche, voté pour Emmanuel Macron contre l'extrême droite, dans l'attente d'une réponse sociale à ce qui s'était exprimé politiquement. pour la troisième fois, nous sommes face à une mobilisation très forte, comme jamais dans ce pays, contre une réforme profondément injuste. De nouveau, vous ne l'entendez pas. Vous jouez avec le feu, c'est extrêmement grave. Cette réforme n'est pas légitime, retirez-la !

! - sont prévus. En effet, à l'article 9, un certain nombre de mesures ont été annoncées, dont le fameux fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle.

le financement du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. Nous prévoyons d'abonder ce fonds à hauteur de 1 milliard d'euros à l'échelle du quinquennat, avec 100 millions cette année et une montée en puissance à hauteur de 200 millions à 250 millions d'euros par an.

par branches, pour les métiers les plus exposés aux troubles musculo-squelettiques. Mme Annie Le Houerou s'est notamment inquiétée de l'équilibre budgétaire et financier de la branche AT-MP.

les décès, notamment dans le secteur des travaux publics et de l'agriculture, de personnes travaillant de manière isolée, qui peuvent être victimes d'un malaise ou subir un accident, par

une priorité. J'aurai l'occasion, dans la loi Travail que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises, de proposer au Parlement des mesures qui permettront d'aller plus loin pour prévenir les accidents graves et mortels. Je le rappelle, nous parlons de 650 morts sur leur lieu de travail et de 1 000 morts au total avec les accidents de trajet et les maladies professionnelles. Mais n'oublions pas

Au fil des débats, nous avons entendu la droite sénatoriale décrire sa vision de la famille. Je ne veux pas être péjorative, mais cette vision me semble tout de même

pour la branche famille, avec le transfert de 2 milliards d'euros des indemnités journalières de la branche assurance maladie vers la branche famille. Alors que les besoins sont urgents, notamment pour la création d'un grand service public de la petite enfance, ces 2 milliards d'euros manqueront, en particulier pour les femmes, les femmes, qui subissent lourdement les conséquences sur leur vie professionnelle de leurs choix familiaux. Je ne peux que regretter et critiquer fortement l'inaction du Gouvernement en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Je suis en colère devant la passivité des pouvoirs publics, qui consiste à accepter d'année en année

pour ne pas subir la décote qui frappe lourdement le montant des pensions de retraite. Au lieu de fixer la durée de travail à 43 ans et l'âge légal à 64 ans, si vous aviez mis en place les mécanismes pour garantir l'égalité salariale, notre système de retraite serait à l'équilibre avec les cotisations supplémentaires, et les pensions des femmes seraient bien supérieures. Permettez-moi de citer Grand Corps Malade : « Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture

et à les accentuer. Six manifestations historiques, 90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, et votre seule réponse est le mépris : mépris envers l'opposition sénatoriale, et surtout mépris du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir, mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime ; retirez-le ! Il y aura encore de grosses manifestations la semaine prochaine, et notamment le 15 mars.

Or, que voyons-nous ? Comme sur les autres sujets, aucune mesure de politique familiale n'accompagne véritablement cette réforme, pour changer l'équation de départ. Ainsi, on entérine

nous devions débattre. Nous avions beaucoup travaillé pour proposer une alternative à vos projets. Nous regrettons d'avoir été bridés, tandis que les Français se sentent privés de la défense de leurs intérêts, ce qui est extrêmement dommageable.

Puis le ministre, qui a manqué une carrière de comique troupier, nous a annoncé dimanche, en grande pompe, qu'il s'agissait d'une réforme de gauche. La vérité, c'est que ce recul de l'âge légal de départ à la retraite répond à un dogme libéral.

l'économiste Michaël Zemmour que vous aimez tant, afin de compenser les baisses d'impôts pour les riches et les entreprises et la baisse des dépenses publiques, qui dégradent nos services publics, pour mieux nous vendre l'efficacité du secteur privé. On l'a moins dit, mais reculer l'âge légal de départ à la retraite, ça sert aussi, en tout cas sur le papier, à garder le marché de l'emploi sous tension. En effet, si on décale l'âge de départ à la retraite, il y aura mécaniquement plus de personnes qui seront contraintes de rester en emploi plus longtemps. la fameuse « réserve » du capital. Si ces personnes restent dans l'emploi, moins de postes se libéreront. La droite sénatoriale veut même organiser la concurrence vers le bas avec les jeunes entrants. Cela soulage le patronat,

90 % des actifs opposés à la retraite à 64 ans, votre seule réponse, c'est le mépris : mépris envers l'opposition sénatoriale, mépris, surtout, du Président de la République

est une réponse attendue pour les aider à faire grandir leurs enfants dans de meilleures conditions. Les professionnels du secteur des métiers de l'enfance et de la protection de l'enfance dénoncent à juste titre un secteur sinistré. L'augmentation du niveau des dépenses de la branche famille pourrait également permettre l'ouverture de places en crèche, le financement d'une vraie réforme du congé parental ou encore la revalorisation des prestations familiales. La parole est

à la maternité et à l'insuffisance d'une politique publique de la petite enfance. Nous avons d'ailleurs dit que les retraites des femmes étaient inférieures de près de 40 % à celles des hommes, et ce ne sont pas les quelques mesurettes que nous avons prises qui y remédieront. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge vient de rendre deux rapports sur l'accueil des enfants de moins de trois ans. Il en ressort que 56 % des parents gardent eux-mêmes leur bébé, faute d'avoir obtenu une place en crèche ou chez une assistante maternelle,

ailleurs, cela a été rappelé, la pauvreté est le quotidien de nombreuses familles. L'inflation pousse toujours plus de familles dans la précarité alimentaire. En témoigne le recours de plus en plus important aux associations de l'aide alimentaire les antennes locales des Restos du Coeur et de la Banque alimentaire de mon département m'ont fait part d'un accroissement très important de leurs bénéficiaires ces derniers mois.

qui concerne les petits, les sans-grade, ceux qui passent, aux yeux de certains bien nés, pour des beaufs ou des ploucs. Eux opposent très concrètement le « quoi qu'il en coûte les dividendes records versés aux actionnaires, les salaires mirobolants, à ce qu'il est « impossible » de faire en matière de retraite, cette prétendue impossibilité

? de la prise en compte des familles pauvres, des familles monoparentales, des enfants nécessitant, dans une perspective républicaine d'égalité, des soutiens adaptés et ciblés en marge et en dehors de l'école ? Ce sujet n'est pas correctement traité dans vos politiques et ne trouve pas de financement dans l'objectif de dépenses de la branche famille. Il faut, comme certaines associations le proposent- je les salue, elles se reconnaîtront -, penser l'action publique en direction des familles et des individus à partir du concept de « pouvoir de vivre

Monsieur le ministre, vous aviez l'occasion de marquer l'histoire de notre pays en allant dans le sens des acquis sociaux, qui font sa fierté, et en donnant de l'espoir à une jeunesse qui aimerait croire que, comme les générations précédentes, sa vie sera meilleure difficile à croire dans le monde instable et fracturé où nous vivons, où les tensions et les guerres se multiplient, difficile, quand nous observons tous les jours l'impact du dérèglement climatique, difficile, dans une France qui voit ses institutions abîmées. Vous aviez, avec cette réforme, la possibilité d'envoyer un signal très fort aux jeunes, aux femmes, à tous ceux qui ont envie de s'investir dans leur travail, de trouver du sens dans leur métier et une motivation au nom de laquelle se dépasser quotidiennement. Au culte du travail pénible, supposé témoigner du sérieux du subordonné, s'oppose l'engagement de travailleurs considérés, heureux dans leur environnement professionnel, mieux formés, dont les perspectives d'évolution de carrière débouchent

ne parle pas des femmes ... Quant aux Français de l'étranger, votre réforme les pénalise doublement : la mobilité, qu'ils ont choisie, les privera de 43 annuités en continu et leur carrière hachée les place de fait dans la catégorie « femmes

proposée ne correspond pas aux aspirations des familles. On nous renvoie à une future loi sur la famille, annoncée depuis longtemps, mais qui a du mal à arriver.

dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. La régression que constitue pour les mères de famille ce projet de réforme a été l'un des fils rouges de nos discussions tout au long de ces derniers jours. Cette régression n'est pas compensée par le dispositif introduit ici même, lors de l'examen du texte par notre assemblée, d'ouverture de la surcote un an avant l'âge légal pour les assurés justifiant de la durée d'assurance requise et bénéficiant des trimestres validés au titre de la maternité.

création d'un service public de la petite enfance, mesure essentielle à l'heure où plus de 200 000 places de crèche seraient nécessaires pour accueillir nos enfants -, cela sans compter, bien sûr, les difficultés supplémentaires qui seront occasionnées par le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Aujourd'hui, 23 millions d'heures de garde hebdomadaires sont assurées par les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, soit l'équivalent de 650 000 emplois à temps plein. Au regard de ces carences, on ne peut que désapprouver les objectifs de dépenses de la branche famille ici présentés, qui sont insuffisants. Voilà un argument de plus pour retirer cette réforme.

présenter l'amendement n° 1772. Pure forme que cet article 17, obligatoire dans un tel texte de financement de la sécurité sociale, et qui concerne la branche famille.

article, obligatoire dans un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, maintient le plafond des dépenses de cette branche au niveau fixé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Si nous proposons la suppression de cet article, c'est parce que les prévisions budgétaires du Gouvernement nous semblent insincères. En effet, elles ne prennent pas en compte les conséquences de cette réforme sur l'ensemble de notre société.

et tous les travailleurs qui auraient eu la mauvaise idée d'exercer un emploi pénible. Reste que les cadres, les emplois de bureau et les professions intellectuelles ne sont pas en reste, puisque tout le monde devra travailler plus longtemps.

d'une violence de classe assez inouïe. La retraite pose la question de la vie et de l'humain ; vous y répondez par de la comptabilité ... Pourtant, il est bien moins coûteux pour la planète et pour notre santé à tous de limiter la place du travail dans nos vies, plutôt que de poursuivre la fuite en avant productiviste que vous défendez. L'histoire retiendra que nous vous avons prévenus avec insistance. Alors que tout le pays défilait encore cet après-midi contre votre réforme des retraites, vous vous êtes inventé une légitimité pour protéger une minorité au détriment de l'intérêt général. Aujourd'hui, nous en sommes à six manifestations historiques 90 % des actifs restent opposés à la retraite à 64 ans. Face à cela, votre seule réponse est le mépris : mépris envers l'opposition sénatoriale et, surtout, mépris du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir, mépris envers les salariés et mépris

avant de concerner la totalité des femmes, ce qui renvoie aux politiques d'égalité professionnelle qui ont été évoquées. Nous aurons aussi l'occasion, dans les prochaines semaines, de donner suite à l'engagement que nous avons pris avec la Première ministre

correspond à une amélioration du niveau de vie, ce qui n'est pas le cas pour les classes moyennes et encore moins pour les classes supérieures. Aussi, quand vous ajoutez deux ans

Le report de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite emportera des conséquences préjudiciables sur la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens, c'est

la sécurité sociale est plus large : ce texte est-il sincère du point de vue de la perte d'autonomie ? Nous pouvons relayer les inquiétudes de la population et des centrales syndicales : dans quel état seront nos concitoyens après avoir dû

vous les travailleurs devront travailler 43 ans jusqu'à 64 ans, vous ne prévoyez aucune mesure pour améliorer le quotidien de nos aînés.

est loin du compte. Après le scandale Orpea, allez-vous continuer à laisser des organismes privés à but lucratif gérer massivement les établissements qui accompagnent nos aînés ? Allez-vous continuer à les laisser faire des profits sur leur dos ? leur dos ? Mettons plutôt à contribution les fonds de pension et les Ehpad lucratifs, qui s'enrichissent sur le dos de nos aînés. J'ai une pensée pour les aides à domicile-

Votre réforme de classe vise à satisfaire les intérêts financiers de l'Union européenne contre les petites gens. Ce débat aura permis de montrer qui sont les défenseurs des intérêts des travailleurs de ce pays.

de mettre à l'ordre du jour de votre politique la fameuse loi Grand Âge, promise depuis très longtemps et toujours repoussée à plus tard.

Je souhaite que votre réponse ne soit plus celle du mépris, le mépris que vous avez signifié à l'encontre de l'opposition sénatoriale, mais, surtout, le mépris du Président de la République envers les syndicats. Votre projet n'est pas légitime. Retirez-le

gouvernement a abandonné cette politique pourtant majeure dans la prise en compte de l'évolution de notre société. Ce manque de souffle, ce manque d'ambition, ce manque d'anticipation entrent en résonance avec une réforme essentiellement financière où le paramétrage est plus important que la réalité sociale.

le contournement parlementaire, la volonté permanente de légiférer en urgence sont des signes qui caractérisent une gouvernance aux abois, soucieuse avant tout de prouver sa capacité à réformer pour combler ses dérives budgétaires et économiques, comme la Cour des comptes, plus particulièrement son président, vient de le confirmer. Aujourd'hui, nous ouvrons un débat qui, sans aucun doute, aura un écho particulier dans les semaines à venir. Votre réforme est avant tout un rendez-vous manqué avec les Français. C'est un rendez-vous manqué avec le Parlement. C'est un rendez-vous manqué avec la démocratie. Vous provoquez les Français. Ils s'en souviendront. Retirez votre réforme, elle n'est pas légitime

pouvant mener à la dépendance. Les moyens dédiés à la branche autonomie prévus à l'article 18 sont ridiculement en deçà des besoins. Nous demandons la suppression de celui-ci comme nous demandons, au nom des Français, le retrait de votre réforme des retraites, injuste et brutale. Les Français étaient d'ailleurs nombreux dans la rue aujourd'hui, pour la sixième journée de mobilisation. Nous savons que 90 % des actifs sont opposés à cette réforme. Cessez ce mépris envers les Français ! Cessez ce mépris envers les parlementaires et demandez au président Macron d'avoir le courage de recevoir les organisations syndicales, qui demandent à le rencontrer ! Retirez votre projet

J'aimerais partager avec vous une information importante : un accord vient d'être trouvé en Espagne pour faire davantage contribuer les hauts revenus au régime de retraite.

présenter l'amendement n° 692. « Les vieillards sont-ils des hommes ? À la manière dont notre société les traite, il est permis d'en douter

Maltraitante institutionnelle, délais d'attente, faible prise en charge : les scandales se multiplient, mais les moyens alloués à l'accompagnement de nos aînés restent insuffisants. Où sont les promesses du président Macron sur l'autonomie ? Nous aurions dû avoir droit à une ambitieuse cinquième branche et à une grande loi sur la dépendance. Dans les faits, la loi a été abandonnée et seules quelques mesures éparses

hausse drastique du taux d'encadrement dans les Ehpad, etc. En 2019, le rapport Libault estimait que la branche autonomie nécessiterait 6 milliards d'euros supplémentaires par an à partir de 2024 et 9 milliards d'euros supplémentaires par an à partir de 2030. L'article 18 de ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale vient corriger à la marge le plafond des dépenses de la branche autonomie pour l'année 2023. C'est une paille au regard des besoins

à un vieillissement démographique sans précédent, alors que le Gouvernement refuse une loi Grand Âge afin de nous préparer collectivement à cette évolution majeure, le budget proposé est insuffisant face aux besoins réels. Vous voulez, de manière dogmatique et obsessionnelle, repousser

Vous tentez d'imposer votre réforme injuste au terme d'un véritable passage en force et au mépris de la mobilisation historique des Français. Travailler jusqu'à l'épuisement, être malade à la retraite

! Nous aurions dû avoir droit à une ambitieuse cinquième branche et à une grande loi sur la dépendance. Rien de tel ! Dans les faits, la loi a été abandonnée et les mesurettes annoncées ont totalement ont totalement disparu. Encore une fois, la branche autonomie n'est pas dotée de moyens suffisants pour faire face aux immenses défis du secteur de l'autonomie, notamment à la crise aiguë dans le recrutement. Nous avons besoin de dizaines de milliers d'embauches et d'une hausse drastique du taux d'encadrement dans les Ehpad. Le rapport de mars 2019 estimait que la branche autonomie nécessiterait 6 milliards d'euros supplémentaires par an à partir de 2024 et 9 milliards d'euros supplémentaires par an à partir de 2030.

l'autonomie, question très importante s'il en est, n'est traitée par votre gouvernement à la hauteur des enjeux ni des difficultés rencontrées par beaucoup de nos compatriotes en perte d'autonomie.

l'amendement n° 1564. L'article 18 prévoit une augmentation de 100 millions d'euros des dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale.

c'est même à des années-lumière des besoins réels et des moyens que nous devrons mobiliser pour faire face au vieillissement de la population. Ce n'est pas avec ces 100 millions d'euros que nous permettrons à chacun de vivre le vieillissement avec sérénité et de profiter d'une retraite en bonne santé, avec une réelle capacité d'autonomie.

est de faire illusion. Il est encore temps de renoncer à cette réforme injuste. Retirez-la ! Au lieu de faire porter les efforts sur ceux qui ont les métiers les plus pénibles, nous pourrions réfléchir collectivement

l'amendement n° 1646. Vous parlez sans cesse du virage domiciliaire. Oui, les Français préfèrent terminer leur vie à domicile. Pour cela, il faut une véritable politique publique et la mise en place d'un service d'aide à la personne digne de ce nom.

Je ne reviendrai pas, mes collègues l'ont fait, sur le scandale des Ehpad privés. La marchandisation de la dépendance est déjà là. Quelle honte !

Selon le baromètre des aidants 2017 de la Fondation April et de BVA, 11 millions d'aidants familiaux, soit un Français sur six, accompagnent au quotidien un proche en situation de dépendance en raison de son âge, d'une maladie ou d'un handicap.

S'ajoutent à cela les disparités sociales liées au métier exercé et ayant des conséquences sur l'usure des individus, mais aussi territoriales au regard de la part que représentent les personnes âgées dans la population des territoires.

les innovations à mettre en oeuvre, à la fois dans l'organisation des services et dans les modalités de prise en charge des personnes dépendantes, doivent être engagés. Les pertes d'autonomie sont progressives et nécessitent une adaptation de leur prise en charge : accompagnement à domicile,

Les moyens qui y sont affectés sont dramatiquement insuffisants ces dernières années. Différents rapports nous ont d'ailleurs alertés sur les grandes problématiques du vieillissement de la population. Tous indiquent deux axes incontournables en la matière d'une part, besoin d'un financement pérenne pour le secteur, d'autre part, nécessité de revaloriser les métiers de l'aide et des soins à domicile. Sur le premier axe, le compte n'y est évidemment pas avec cet article ; quant au second,

Emmanuel Macron avait annoncé une réforme Grand Âge et autonomie pour avant l'automne 2019. Des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap, leurs familles et les associations l'attendaient avec beaucoup d'espoir, de même que les personnels qui les accompagnent. Il n'y a pas eu de réforme ; il n'y a eu que du mépris, le même mépris que celui qui a été opposé aujourd'hui aux 90 % d'actifs qui sont opposés à cette réforme injuste, le même mépris que celui qui est opposé aux millions de personnes qui ont participé aux six manifestations historiques que nous venons de connaître, le même mépris que celui que vous opposez à l'opposition sénatoriale depuis le début de ces débats. par le mépris jupitérien du Président de la République envers les syndicats et les organisations de jeunesse qu'il refuse de recevoir. Afficher tant de mépris ne vous donne pas plus de légitimité, bien au contraire. Retirez ce projet et occupez-vous des vraies urgences.

En 2050, selon l'Insee, 4 millions de seniors seront en situation de perte d'autonomie. Vous n'y répondez pas.

je vous rappellerai maintenant l'essentiel : six journées de manifestations d'ampleur considérable, l'immense majorité des actifs opposés à la retraite à 64

Aucune réforme, si nécessaire soit-elle, ne peut être menée à bien sans une large adhésion de toutes les parties intéressées [ ...] Il apparaît clairement que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les manifestations en cours [ ...] en sont la preuve. j'ai décidé de retirer l'actuel projet de loi. » Ce sont les mots du président Jacques Chirac, le 8 décembre 1986. Puisse le président Emmanuel Macron faire preuve d'un même sens de la cohésion nationale. Ce projet n'est pas légitime. Il faut le retirer

que vous prévoyez pour la branche autonomie de la sécurité sociale. J'en profite pour vous dire combien votre réforme est regrettable pour tous les corps qu'elle va abîmer, casser, les maladies professionnelles qu'elle va déclencher en nombre, les décès prématurés qu'elle va provoquer. En repoussant l'âge de départ à la retraite à 64 ans, en ajoutant des années de cotisation à toutes celles et à tous ceux qui travaillent, porter le nombre à 43 ans et 44 ans, vous avez fait le choix de faire payer le travail pour protéger le capital, à qui vous ne demandez rien. Les profits des entreprises, les dividendes ne sont pas égratignés. Au contraire, ils sont concentrés et renforcés. Demander aux Français de travailler plus longtemps parce qu'ils vivraient plus longtemps est une imposture, d'autant que, vous le savez bien, l'espérance de vie, comme celle d'une retraite en bonne santé, varie selon la classe sociale et l'emploi occupé.

actifs opposés à la retraite à 64 ans, votre seule réponse, c'est le mépris : mépris envers l'opposition sénatoriale, mépris, surtout, du Président de la République envers les syndicats, qu'il refuse de recevoir, mépris envers les salariés et les Français. Votre projet n'est pas légitime. Retirez-le !

44.3, ... 53-10 ! ... article 38, article 42, 62 à 64 ans, déficit à 3 % présenté comme un dogme. Vous aimez les chiffres, on peut le dire, surtout quand ils vous arrangent. Vous aimez les chiffres quand ils profitent aux plus riches. Vous aimez les chiffres quand il s'agit de milliards d'euros pour quelques-uns. Vous aimez les chiffres, parce que, tout simplement, vous n'aimez pas les gens. 11 millions de personnes pauvres en France- la moitié sont des femmes -et 17 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Oui, derrière ces chiffres, il y a des gens, des vies. gens, des vies. Votre réforme va aggraver encore plus la vie des plus pauvres. À 64 ans, un tiers des plus pauvres, c'est-à-dire un tiers de ceux qui ont les métiers les plus difficiles, sont déjà morts. Ils auront cotisé pourtant toute une vie pour payer la retraite des générations précédentes. Cette réforme retire tout simplement de la vie aux plus pauvres. Elle institutionnalise l'injustice. Les plus riches pourront échapper à votre réforme, les pauvres, non. Votre réforme va précariser les plus âgés et les plus pauvres, et pénaliser les jeunes et les femmes. c'est le nombre de manifestations historiques dans le pays ; un million, le nombre de signataires, aujourd'hui, pour une consultation citoyenne ; 90 %, c'est le pourcentage d'actifs contre votre réforme. Pour une fois, s'il vous plaît, écoutez les gens, écoutez ces gens-là. Retirez votre réforme